L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports

Mme la rapporteure. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis que nous puissions examiner aujourd’hui les conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports, que le Sénat a adoptée il y a un an. Il s’agit, je le crois, d’un texte profondément utile, qui permet d’apporter des réponses concrètes et opérationnelles à une problématique bien réelle. Selon une enquête publiée récemment par le ministère de l’intérieur, 40 % des Français déclareraient se sentir en insécurité dans les transports. Difficile de leur donner tort, quand on sait que près de 120 000 faits de vols et de violences y ont été commis au cours de la seule année 2023. Les gares ferroviaires, les stations de métro et de bus, les réseaux ferrés ainsi que les véhicules de transport sont, par nature, vulnérables à certaines menaces – je pense en particulier à la menace terroriste et aux violences sexistes et sexuelles. Il est de notre responsabilité

Dans le même temps, il nous appartenait de veiller à préserver, d’une part, les droits et libertés constitutionnels et, d’autre part, la cohérence du continuum de sécurité dans lequel les services de sûreté de la SNCF et de la RATP s’inscrivent parfaitement. Le texte de compromis qui résulte des travaux de la commission mixte paritaire reflète fidèlement les préoccupations des deux assemblées, tout en apportant les garanties nécessaires pour assurer sa sécurité juridique et son opérationnalité. Je me concentrerai sur quelques points essentiels. Les articles 1 à 3 permettent une extension significative des prérogatives des agents des services internes de sécurité de la SNCF – la des réseaux (GPSR). Le texte assouplit les conditions dans lesquelles ils peuvent procéder à des palpations de sécurité et leur donne de nouvelles facultés en matière d’interdiction d’entrée dans les gares, de saisie d’objets dangereux et d’intervention sur la voie publique. Ces mesures, adoptées par le Sénat, sont confortées, sous réserve d’ajustements que nous avons jugés nécessaires pour assurer la constitutionnalité du dispositif de saisie. Le texte prend également en compte les enjeux de sûreté liés à l’ouverture à la concurrence des transports, qui implique l’arrivée d’opérateurs ne ne disposant ni de Suge ni de GPSR. C’est la raison pour laquelle l’article 7 permet l’accès d’agents d’Île de France Mobilités au centre de coordination opérationnelle de sécurité L’article 2 , introduit par l’Assemblée nationale, permet de renforcer les prérogatives des agents de sécurité privée en matière d’éviction des véhicules dans les gares. Le texte issu de la commission mixte paritaire conserve les dispositions permettant de renforcer les moyens technologiques des opérateurs de transports, prévues aux articles 8 à 11. Il conserve ainsi la pérennisation du recours aux caméras piétons

part, sur le recours aux caméras embarquées dans les bus scolaires à Mayotte, qui sont malheureusement la cible d’attaques récurrentes,

ces dispositifs, il nous est apparu que certaines garanties supplémentaires devaient être apportées, en particulier concernant la captation du son, afin d’assurer leur sécurité juridique. La proposition de loi renforce également l’arsenal pénal de la police des transports. L’article 14 aggrave la répression des oublis et abandons de bagages, qui sont lourds de conséquences

: le et. Ce texte, d’initiative sénatoriale, intègre enfin des mesures importantes issues des travaux de notre assemblée. L’article 13 institue ainsi une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les réseaux de transport, dispositif qui a déjà été voté à deux reprises par le Sénat.

Monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est avec plaisir que je représente aujourd’hui mon collègue Philippe Tabarot, ministre chargé des transports, retenu par des négociations européennes, pour la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi relative au au renforcement de la sûreté dans les transports, un texte qui s’est fait attendre, mais dont l’examen parvient aujourd’hui à son terme ! Ce texte revêt une symbolique toute particulière, puisqu’il revient dans cet hémicycle

Le Gouvernement y voit une preuve de plus, s’il en fallait, que la Haute Assemblée produit de grands textes, mais favorise aussi les destinées de ceux qui les promeuvent ! On peut en effet se poser la question ! J’en profite d’ailleurs pour saluer la qualité du travail réalisé par votre assemblée sur ce texte. Je remercie tout particulièrement la rapporteure Nadine Bellurot, la présidente de la commission des lois Muriel Jourda, les membres de la commission mixte paritaire, ainsi que l’ensemble des sénatrices et sénateurs ayant contribué à cette proposition de loi. Avant toute chose, je tiens à rappeler que cette démarche s’inscrit dans la continuité du travail précurseur engagé par les députés socialistes Gilles Savary et Bruno Le Roux en 2016, qui ont posé les premiers jalons d’une politique ambitieuse de sécurité dans les transports. Cela démontre que la sûreté n’est ni de droite, ni du centre, ni de gauche : c’est une exigence républicaine qui nous rassemble tous. Le texte que nous examinons aujourd’hui s’inscrit dans cette même approche consensuelle, enrichie par le travail conjoint des deux assemblées. Il répond avant tout à une réalité préoccupante : 110 000 personnes victimes de vols, violences ou escroqueries dans nos transports en 2024, une augmentation de 15 % des violences sexuelles et sexistes au cours de la seule année 2023, des agressions contre les agents qui ne cessent de croître. Face à ces défis, nous ne pouvions rester immobiles. La commission mixte paritaire qui s’est réunie le 6 mars dernier est parvenue à un accord équilibré qui préserve l’esprit initial du texte tout en l’enrichissant de manière substantielle. Permettez moi d’en détailler les principales avancées. Tout d’abord, nous renforçons significativement les moyens d’action des services de sûreté. Les agents de la Suge et du GPSR pourront désormais procéder à des palpations de sécurité sans autorisation préalable du préfet lorsque des éléments objectifs l’exigent. Ils pourront également saisir les objets dangereux, une mesure particulièrement attendue par les opérateurs. Le texte leur accorde également un droit de poursuite sur la voie publique, lorsque le caractère inopiné ou urgent de la situation le justifie. vise avant tout à renforcer notre continuum de sécurité entre les forces de polices nationale et municipale, les agents de la Suge et du GPSR, et les agents de sécurité privée. a également maintenu des dispositions essentielles concernant les interdictions d’accès aux transports pour les auteurs d’infractions graves, tout en prévoyant des garanties importantes.

La lutte contre les bagages abandonnés, qui paralysent trop souvent nos réseaux, fait l’objet d’un dispositif gradué de sanctions. Le texte permet désormais aux opérateurs de déposer plainte pour le compte de leurs agents victimes d’agressions, avec leur accord. Il renforce également le dispositif Stop fraude lancé au début du mois de janvier 2025. Outre les mesures adoptées, ce texte aura également permis d’engager un travail sur les dispositifs actuels. Le Gouvernement a lancé avec les opérateurs, la direction de la sécurité routière et l’Imprimerie nationale un travail visant à améliorer le dispositif Vérif permis, qui permet aux opérateurs de bus de vérifier la validité des permis de conduire de leurs conducteurs. Ce texte Ce texte vise également à anticiper les enjeux de l’ouverture à la concurrence en prévoyant la remise d’un rapport d’évaluation sur les conséquences en matière de sûreté. Le Gouvernement, qui est en général peu adepte des rapports, soutient cette disposition, car il est impératif de réfléchir à notre modèle de demain. La proposition de loi apporte des réponses concrètes et pragmatiques aux défis de la sûreté dans nos transports, sans jamais perdre de vue l’équilibre nécessaire entre sécurité et libertés. En effet, il s’agit non de restreindre les libertés, mais bien au contraire de garantir la première d’entre elles, celle d’aller et venir sereinement. Je sais cette assemblée particulièrement attachée à la sécurité du quotidien de nos concitoyens. Le texte qui vous est soumis aujourd’hui est fidèle à l’esprit qui a présidé à sa conception : pragmatique, équilibré, il est résolument tourné vers l’efficacité. Il démontre que, lorsque la représentation nationale travaille dans un esprit constructif, elle est capable de produire des avancées majeures pour nos concitoyens. les sénateurs, je vous invite donc à adopter les conclusions de la commission mixte paritaire sur cette proposition de loi qui, à coup sûr, marquera une nouvelle étape importante dans notre politique de sûreté

Chercher à favoriser des déplacements sûrs, tenter de renforcer la sérénité dans nos transports publics, les transports scolaires ou lors des périodes de vacances est un impératif pour les élus que nous sommes. Néanmoins, avant toute chose, il me semble judicieux de rappeler, au moment où nous sommes invités à voter sur des dispositions qui ont fait l’objet d’un accord en commission mixte paritaire, que nous allons nous prononcer sur une proposition de loi déposée par un sénateur des Alpes Maritimes, M. Philippe Tabarot,

n’hésitant jamais à dénigrer la représentation nationale. Lors des différentes discussions qui ont accompagné l’élaboration du texte, le groupe du RDSE a rappelé, à de nombreuses reprises, la nécessité d’assurer un continuum de sécurité pour les usagers et de le faire en facilitant le travail des agents des différents services qui en ont la charge. L’an dernier, en accord avec le promoteur de ce texte et bon nombre d’observateurs, décideurs, acteurs associatifs ou agents des réseaux de la SNCF ou de la RATP, nous avons souligné notre inquiétude face à la dureté de certains chiffres.

de dix ans, et 91 % des victimes étaient des femmes ! Comment accepter sans ciller de tels constats ? À l’évidence, il était nécessaire, que dis je, il était indispensable, pour commencer à y répondre, pour commencer à y répondre, d’octroyer aux agents les moyens nécessaires à la sécurisation des transports en commun. Parallèlement, il était urgent de combler les lacunes de la législation pénale en vigueur. Toutefois, et chacun ici s’en souvient, nous avons formulé plus que des réserves devant certains amendements dont l’adoption aurait remis en cause l’équilibre entre sécurité et libertés publiques. Je constate, et le groupe du RDSE fait de même, que la commission mixte paritaire a su maintenir un juste équilibre dans ses conclusions. Sans doute ce résultat a t il été possible parce que le pragmatisme l’a emporté. Ainsi, le niveau des amendes relatives aux oublis de bagages, qui empoisonnent le quotidien des usagers des gares et occasionnent des retards horripilants, a été établi de façon raisonnable. Nous remarquons avec satisfaction que le texte issu du dialogue constructif entre députés et sénateurs clarifie les missions des services de la SNCF et de la RATP, tout en renforçant leurs pouvoirs sur le terrain. Par ailleurs, les dispositions de vidéosurveillance algorithmique ou liée à l’intelligence artificielle, expérimentées durant les jeux Olympiques de 2024, seront prolongées jusqu’en 2027. Nous souhaitons que ce délai permette d’établir les évaluations indispensables pour juger de leur efficacité et décider de leur pérennisation, sans remise en cause des droits fondamentaux des personnes. À l’évidence, ce texte apporte des réponses concrètes afin de favoriser une vision plus globale de la sécurité, de mieux se déplacer et de voyager plus sereinement. Ne nous leurrons pas, cependant. Le chantier pour restaurer pour restaurer la sécurité dans les transports publics ne s’arrête pas à la porte des gares et ne se limite pas aux rames de métro ou de chemins de fer, pas plus qu’aux bus qui sillonnent nos villes et nos campagnes. Personne ne peut ignorer la prégnance de la menace terroriste ni la réalité des actes délictueux et des incivilités qui émaillent la vie quotidienne des Français. Il nous appartient, en tant que législateurs, de continuer à forger des réponses concrètes, pratiques, qui ne cèdent pas à l’idéologie, mais qui privilégient le pragmatisme pour continuer, chaque jour, à améliorer la vie de nos concitoyens. Cette tâche est une invitation collective à renforcer l’éducation, recoudre le lien social et à veiller à l’application de mesures justes, mais fermes, pour lutter contre les incivilités et les violences. C’est un combat de longue haleine. Ce texte y participe. C’est pour cette raison, mes chers collègues, que le groupe du RDSE votera pour son adoption.

que je salue, ce texte s’inscrit dans une continuité juridique et répond malheureusement à une augmentation de la violence et des actes d’incivisme dans notre société.

Nous examinons donc aujourd’hui le texte approuvé par la commission mixte paritaire le 6 mars dernier, quasiment jour pour jour à la date anniversaire de la promulgation Cette coïncidence a été rendue possible grâce non seulement au travail de qualité réalisé par les deux rapporteurs, notre collègue Nadine Bellurot et le député Guillaume Gouffier Valente, que je salue également, lesquels ont su lever des objections et parvenir à un accord sur les trente deux articles constituant ce texte, mais aussi à une volonté de dialogue de l’Assemblée nationale et du Sénat ayant permis de supprimer des dispositions qui auraient pu être déclarées anticonstitutionnelles. Je pense à la possibilité de transaction en en cas de délit. Ce travail de consensus a répondu aussi au principe, maintes fois répété par le Conseil d’État, du juste équilibre entre sécurité et préservation des libertés, précepte essentiel pour préserver notre État de droit.

Comme il a été rappelé, le nombre annuel total de faits de vol et de violence recensés dans les transports s’est élevé à 118 440 en 2023. Chaque année, depuis 2016, cette statistique

et l’augmentation de moyens humains dans les transports publics. Je suis persuadée qu’il continuera à baisser grâce aux nouvelles prérogatives attribuées aux agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP et aux nouveaux de la RATP et aux nouveaux moyens technologiques accordés à ces opérateurs de transport par le présent texte, telle la pérennisation du recours aux caméras piétons. Face à ces nouveaux droits, je tiens aussi à relever que le texte crée de nouvelles obligations aux transporteurs, comme celle d’interdire la fonction de conducteur de transport de véhicule aux personnes mentionnées au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. Il prend aussi en compte le traitement de nouvelles formes d’incivilités par la création notamment du délit de. Mes chers collègues, au regard de l’esprit consensuel qui a présidé à l’élaboration de ce texte, je n’en dirai pas plus, si ce n’est que le groupe Union

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, il y a un peu plus d’un an, le Sénat adoptait la proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports, déposée par le sénateur Philippe Tabarot, aujourd’hui ministre. Déjà, à l’époque, le groupe CRCE K s’était opposé à ce texte, pour toutes les incohérences qu’on y trouve et l’ensemble des sanctions proposées, des plus inefficaces aux plus disproportionnées. Son passage à l’Assemblée nationale, puis en commission mixte paritaire, n’a pas suffi à lever nos interrogations. Jugez plutôt. On crée un délit de, qui est le fait d’« utiliser comme engin de remorquage ou de se tenir sur les marchepieds ou à l’extérieur dudit véhicule pendant la marche sans autorisation ». C’est en effet un geste stupide, dangereux certainement, dont la sanction sera suffisamment douloureuse en cas de choc pour que celui qui en sera l’auteur ne recommence pas. C’est toutefois suffisamment rare pour que, je pense, personne ici n’y ait jamais été confronté. Nous nous réjouissons évidemment de la suppression du délit d’incivilité d’habitude, de la suppression du traitement algorithmique pour accélérer les réquisitions judiciaires, ainsi que de toutes les mesures qui, nous n’en doutons pas, seraient certainement plébiscitées dans d’autres pays. Malheureusement, il en reste d’autres. Je pense au renforcement des sanctions à l’égard des oublis de bagages, alors que ces oublis sont, par définition, non intentionnels, au renforcement des prérogatives des agents de police judiciaire adjoints dans les transports, là où ce n’est pas forcément leur rôle, et à la possibilité d’intervenir dans l’espace public, en dehors des gares, pour les agents de sûreté, y compris d’entreprises privées.

Quels trains allez vous sécuriser, lorsque toutes les petites lignes auront fermé ? Quels passagers aurez vous à protéger, lorsqu’ils seront tous dans leur voiture ou bloqués dans leur village où la gare aura fermé ?

L’ouverture à la concurrence incitera les opérateurs à se concentrer sur les lignes les plus rentables et à délaisser les moins empruntées, qui sont pourtant les plus indispensables pour désenclaver nos territoires, et encourager leur dynamisme et la transition des mobilités. sont valables pour le transport de voyageurs, mais aussi pour le transport de marchandises. Les deux sont mis à mal. Alors qu’il faudrait légiférer pour soutenir le développement et l’entretien du réseau, alors qu’il faudrait parler service public des transports, nous parlons et caméras de surveillance Il est plus facile de taguer un train à l’arrêt qu’un train qui roule, et moins anxiogène d’attendre dans une gare des trains aux fréquences régulières, plutôt qu’un train aux passages aléatoires, retardés ou annulés. Oui, il faut renforcer la sûreté des transports, et d’abord en rénovant les voies ferrées pour éviter les accidents, mais aussi pour ne pas avoir à ralentir, à perdre en compétitivité et à devoir finalement fermer lignes. Vous l’aurez compris, le groupe CRCE K votera contre ce texte, en espérant que le ministre chargé des transports profitera de ses nouvelles fonctions pour présenter des projets de loi plus audacieux et utiles

Monsieur le président, monsieur le ministre,

Nous saluons les travaux et la plupart des constats et diagnostics de l’auteur de la proposition de loi et de la commission. Cependant, comme toujours, nous déplorons qu’aucune mesure d’évaluation des mesures existantes n’ait été réalisée au préalable. Le texte adopté par la commission mixte paritaire ne tient pas suffisamment compte des écueils que nous avions relevés dès la lecture de ce texte dans notre hémicycle. Commençons par le désengagement progressif de l’État en matière de sécurité publique, qui est sa compétence régalienne. Le sujet est pour nous crucial : ce transfert, ces délégations de compétence, ce continuum de sécurité, deviennent trop souvent un continuum sécuritaire. Mon collègue Thomas Dossus a déjà défendu cette position lors de l’examen de ce qui allait

qui prévoit l’extension du continuum de sécurité – à savoir cette confusion de compétences entre les différentes forces de sécurité –, avec le libre accès des agents de la police municipale aux espaces et matériels roulants des transports de voyageurs, aux espaces de transport et aux trains en circulation.

la confiance des usagers envers les agents. Ce texte a pour ambition d’accroître les prérogatives des forces de sécurité dans les transports en commun, les gares et leurs abords, mais il crée aussi de nouveaux délits et renforce massivement les dispositifs de surveillance dans l’espace public.

l’article 19, nous avions fait part, dès la première lecture en séance publique, de notre opposition à un décret qui fixerait les modalités de sélection des personnes morales de droit privé amenées à récolter des données sensibles, fiscales et sociales auprès des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale dans les cas de recouvrement des sommes dues pour des contraventions.

Pour autant, les mesures prévues dans ce texte ne permettent que trop peu la prévention de délits ou d’attaques, et font peser sur les utilisateurs ou usagers le risque d’un contrôle arbitraire au delà du raisonnable.

d’avoir une approche globale de la sûreté dans les transports. Il s’agit, en quelque sorte, d’une occasion manquée. Néanmoins, certaines dispositions sont intéressantes et nous y sommes favorables.

la période des jeux Olympiques nous a fait découvrir un Paris quelque peu idéalisé : une ville propre, des transports en commun fonctionnels, et surtout une tranquillité publique que la capitale n’avait pas connue depuis des décennies. Cet épisode enchanté n’aura malheureusement duré qu’un été et concerné que quelques villes de France. L’utopie d’une ville parfaite dans une société

constamment en retard et peu sûrs. Nos collectivités territoriales sont le fer de lance du développement des transports en commun. Elles investissent constamment pour que les trains, les trams ou les métros soient plus nombreux, plus propres et ponctuels. Cependant, pour convaincre nos concitoyens d’emprunter ces transports et récompenser les investissements des élus locaux, la question de la sûreté doit impérativement être résolue par les opérateurs et, surtout, par les services de l’État.

la très nette augmentation des incivilités et des violences, et plus particulièrement des violences sexuelles, doit nous alerter. Nous devons nous adresser aux 3 374 victimes de violences sexuelles dans les transports en commun enregistrées

prévoit notamment un droit de poursuite sur la voie publique, un pouvoir d’éviction des transports en commun et la possibilité de prononcer une interdiction d’accès à ces transports. La capacité des agents de visionner les images de vidéosurveillance captées dans les transports pour identifier les auteurs d’infractions sera étendue, et une expérimentation leur permettra d’être équipés de caméras piétons. Pour mieux protéger nos enfants, les opérateurs de transport scolaire à Mayotte auront la possibilité de filmer la voie publique au moyen de caméras frontales et latérales embarquées. Pour réagir aux situations les plus violentes, certains agents chargés de la sécurité des voyageurs pourront même être équipés de pistolets à impulsion électrique.

Monsieur le président, monsieur le ministre,

l’ai évoqué dans mon intervention en discussion générale lors de l’examen en séance publique le 13 février 2024, cette proposition de loi répond – j’en suis convaincu – à une demande forte de nos concitoyens, mais aussi de nos opérateurs de transport et de ceux qui y travaillent au quotidien, dans des conditions que nous savons parfois difficiles et violentes. Quelque 2 407 victimes de violences sexistes et sexuelles et sexuelles ont ainsi été comptabilisées en 2023, dont 62 % en Île de France. Parallèlement, ainsi que le relève la SNCF sur son réseau, on observe une croissance exponentielle du nombre d’objets dangereux,

Le texte institue tout d’abord un droit de poursuite au bénéfice des agents de sûreté de la SNCF et de la RATP lorsqu’un contrevenant se rend sur la voie publique après avoir commis une infraction à l’intérieur d’une emprise ou d’un véhicule. Il pérennise par ailleurs l’expérimentation, qui a pris fin le 1 octobre dernier, prévoyant le port de caméras piétons pour les contrôleurs et pour l’ensemble des agents des services internes de sécurité. Il s’agit de pérenniser « un moyen plébiscité par les agents pour diminuer les tensions en cas d’agression », a fait valoir le ministre chargé des transports Philippe Tabarot, qui – preuve de sa ténacité sur le sujet – s’est rendu

de loi autorise, à titre expérimental également, les conducteurs d’autobus et d’autocars à déclencher, en cas de danger, un système de captation sonore auquel pourrait accéder en temps réel le poste de contrôle et de commandement. Conformément aux souhaits du Sénat, le texte élargit par ailleurs les prérogatives des forces de sécurité dans les transports – sûreté ferroviaire pour la SNCF, GPSR pour la RATP qui pourront procéder à des palpations sans avoir besoin du feu vert du préfet lorsqu’il existe des éléments objectifs laissant penser qu’une personne pourrait détenir des objets susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des voyageurs. Ils pourront en outre intervenir aux abords des gares et saisir des objets considérés comme potentiellement dangereux. La proposition de loi crée une nouvelle interdiction d’entrée en gare, qui vise les personnes dont le comportement au seuil d’une emprise trouble l’ordre public et pourrait compromettre la sécurité des personnes ou la régularité des circulations, ainsi que celles qui refusent une inspection visuelle, la fouille de bagages ou des palpations de sécurité. Ces avancées sont majeures. Le texte impose également à l’ensemble des entreprises ferroviaires de mettre en place un numéro d’appel unique pour permettre aux voyageurs de signaler rapidement des situations qui présentent un risque pour leur sécurité ou celle des autres voyageurs.

Cet algorithme analyse les images de vidéosurveillance afin de repérer des comportements suspects. Nous devons garder une chose en tête : la plus grande des restrictions de libertés, c’est lorsque nos concitoyens renoncent à utiliser les transports en commun à certaines plages horaires ou sur certaines lignes. À nous de leur faire aimer les transports en commun ! En définitive, ainsi que l’avait résumé Jean Pierre Farandou lors de son audition au Sénat, cette proposition de loi contribue à apporter un « supplément d’efficacité dans l’action ». C’est la raison pour laquelle le groupe Les Républicains votera le texte issu des travaux de la commission mixte

Un chiffre glaçant publié récemment nous rappelle la nécessité d’agir : en 2024, nos services de police et de gendarmerie ont enregistré près de 3 400 victimes de violences sexuelles dans les transports en commun,

Nous partageons pleinement sa volonté. Sans suspense, mon groupe votera unanimement en faveur des conclusions qui nous sont présentées aujourd’hui, plus d’un an après l’adoption du texte en première lecture au Sénat.

pouvoir circuler plus librement et plus sûrement dans les lieux de transport public. En cas d’adoption définitive – ce dont je ne doute pas –, il sera possible, pour les pour les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, de procéder à des palpations de sécurité sans autorisation préalable du préfet, dans certaines situations

Concernant l’article 2 et l’intervention de ces agents sur la voie publique, un compromis a, là encore, été trouvé. Alors que la possibilité de doter les agents du service interne de sécurité de la SNCF de pistolets à impulsion électrique a été conservée, la commission mixte paritaire a écarté l’alignement des règles d’usage des armes des agents de la Suge et du GPSR sur celles des policiers et des gendarmes, tout en leur permettant de bénéficier du cadre relatif à la « légitime défense élargie » et au « périple meurtrier

de la mobilité (AOM) pour déterminer les conditions dans lesquelles les agents de la police municipale ou les gardes champêtres pourront accéder aux espaces de transport.

Ainsi, pendant trois ans, les opérateurs de transport scolaire à Mayotte pourront filmer la voie publique au moyen de caméras frontales et latérales embarquées, de même que les opérateurs de transports guidés urbains seront autorisés à installer des caméras frontales embarquées sur les matériels roulants. Pour deux ans, la captation et la transmission du son dans les bus et les cars à des fins de sécurité des conducteurs sont rendues possibles dans certaines conditions. Quant à l’expérimentation de traitements algorithmiques sur les images de vidéosurveillance dans le cadre de manifestations sportives, récréatives ou culturelles, elle sera encore possible jusqu’au 1 mars 2027. À l’inverse, l’article 9, qui encadrait l’utilisation à titre expérimental de traitements algorithmiques sur des images issues des caméras de la SNCF et de la RATP en temps différé, a été supprimé. Au volet des sanctions,

Il sera nécessaire d’en faire une publicité large à destination des voyageurs. Le délit de, prévu par la proposition de loi, pourra quant à lui être sanctionné de 3 750 euros d’amende. Enfin, mon groupe se félicite que l’exploitant d’un réseau de transport public puisse bientôt déposer déposer plainte pour le compte de ses agents victimes d’atteinte volontaire à leur intégrité physique ou psychique, de menaces, d’actes d’intimidation ou d’outrage, et que toute personne définitivement condamnée pour des infractions violentes ou sexuelles, ou pour une infraction à caractère terroriste, soit interdite d’exercer comme conducteur ou d’intervenir

L’ordre du jour appelle le débat préalable à la réunion du Conseil européen des 20 et 21 mars 2025, organisé à la demande de la commission des affaires européennes. Je vous rappelle que, dans ce débat, le Gouvernement aura la faculté, s’il le juge nécessaire, de prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes l’orateur disposera alors à son tour du droit de répartie, pour une minute. Monsieur le ministre délégué, vous pourrez donc, si vous le souhaitez, répondre après chaque orateur, une fois que celui ci aura retrouvé une place dans l’hémicycle.

Nous devons désormais rester plus unis et mobilisés que jamais, en ce moment décisif où les États Unis souhaitent accélérer les négociations de paix et où Moscou accentue sa pression militaire sur les troupes de Kiev dans la région de Koursk. Sur le fond, nous sommes d’accord sur cinq points fondamentaux. ne doit avoir lieu sans l’Ukraine. Aucune négociation sur la sécurité européenne ne doit être menée sans les Européens. Toute trêve ou tout cessez le feu doit avoir lieu dans le cadre du processus menant à un accord de paix global. Tout accord de paix doit s’accompagner de garanties de sécurité robustes et crédibles pour l’Ukraine.

Nous devons travailler, avec les Européens, à des garanties de sécurité robustes et crédibles. Sur ce point, le Président de la République a, encore une fois, donné l’impulsion, en invitant la semaine dernière tous les chefs d’état major des armées de nos partenaires à Paris, pour étudier l’ensemble des options envisageables. Cela suppose également de maintenir un soutien solide à l’Ukraine, en accélérant notamment le déboursement de notre prêt et en veillant à ce qu’il profite en priorité aux industriels européens. Nous continuerons à avancer sur ces deux volets jeudi et vendredi, avec nos partenaires européens.

de la guerre d’agression russe en Ukraine et l’adoption de l’agenda de Versailles durant la présidence française, après le diagnostic établi par le rapport Draghi, après les prises de position de la nouvelle administration américaine et

Ce changement d’échelle, nous l’avons acté le 6 mars dernier. Nous nous sommes mis d’accord, pour la première fois, sur une liste de domaines prioritaires dans lesquels nous devons investir ensemble, en tant qu’Européens, et sur des options de financement à explorer, à partir notamment des propositions de la présidente de la Commission, dans le cadre du plan ReArm Il faut aller maintenant le plus vite possible dans la mise en œuvre. Nous attendons les premières propositions de la Commission, qui auront lieu dès mercredi, lors de la publication d’un livre blanc sur la défense et d’un paquet législatif qui concrétisera les options de financement.

bien sûr de la pression des événements et du discours de l’administration américaine. Une Europe forte et indépendante est aussi une Europe prospère, capable d’innover et d’assurer sa production dans les domaines les plus stratégiques. Nous aurons ainsi, lors du Conseil européen, un nouvel échange sur la compétitivité. Discours de la Sorbonne, agenda franco allemand de Meseberg, rapports Letta et Draghi, agenda stratégique européen, déclarations de Versailles, Grenade et Budapest : nous n’avons eu de cesse d’appeler à un sursaut européen. La boussole pour la compétitivité et le pacte pour une industrie verte, récemment présenté par la Commission, témoignent que notre ambition en la matière est partagée par les institutions européennes. Il faut désormais que les propositions se concrétisent et qu’elles produisent leurs effets rapidement. Nous accélérons aussi la mise en œuvre de l’agenda de simplification,

notamment en direction de nos PME. Celles ci devraient voir leurs charges administratives allégées. Nous pensons toutefois que cette démarche doit aller plus loin, notamment pour simplifier la vie de nos agriculteurs, comme le Président de la République le comme vous le savez, il ne suffit pas de définir un agenda industriel ambitieux : sa mise en œuvre peut, à tout moment, être compromise par des menaces ou des actions unilatérales, susceptibles d’exercer des effets préjudiciables graves sur nos économies et nos entreprises. Nous devons donc assurer notre sécurité économique et, dans un monde de plus en plus fragmenté, nous défendre collectivement à la fois contre la concurrence déloyale, les surcapacités et les décisions tarifaires hostiles.

Alors que l’alimentation pourrait devenir, dans le contexte d’exacerbation des tensions géopolitiques, une arme utilisée par des puissances rivales, telles que la Russie, efficacement à ces enjeux, nous doter d’un agenda pour renforcer la souveraineté alimentaire européenne, en garantissant la capacité productive de l’Union, en préservant les revenus des agriculteurs, en établissant

Nous serons également vigilants sur la politique de cohésion : nous devons préserver les intérêts de nos régions, notamment ultrapériphériques. Cet effort d’investissement massif que nous souhaitons ne sera possible que si nous trouvons de nouvelles sources de financement du budget européen.

Une Europe forte, c’est aussi une Europe qui prouve à ses citoyens qu’elle est capable d’agir efficacement face aux défis qui les touchent. Je pense en particulier à la question de la maîtrise de l’immigration. Les chefs d’État et de gouvernement feront notamment le point sur la mise en œuvre – c’est et l’asile, qui nous dote de nouveaux outils indispensables pour assurer le contrôle de nos frontières. Il est également primordial de faciliter les éloignements et les expulsions. La Commission a proposé une nouvelle législation, afin de faciliter les retours.

dans un ordre mondial en plein bouleversement, une Europe forte est une Europe capable d’avoir une action extérieure stable, lisible et cohérente pour nos partenaires, face à une administration américaine plus que jamais imprévisible. Cela concerne notamment notre action au Proche Orient, qui sera également à l’ordre du jour du Conseil européen. Au Liban, nous devons accompagner la dynamique de changement engagée par le renouvellement de l’exécutif et continuer à soutenir la construction d’une paix durable dans le sud. La France continuera à jouer dans ce processus le rôle clé qu’elle a joué ces derniers mois. En Israël et dans les territoires palestiniens, il nous importe de tout faire pour préserver le cessez le feu et la perspective d’une solution à deux États, face à l’imprévisibilité de l’action américaine, en soutenant unanimement le plan arabe pour Gaza.

inclusivité et représentativité dans le processus ; respect des droits humains ; respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Syrie ; et mise en œuvre d’une action ferme en matière de lutte antiterroriste. Nous devons être très clairs sur ce point : notre engagement, notamment en ce qui concerne la levée des sanctions, est réversible. un dernier mot sur notre action en faveur de l’océan. L’Europe doit être au rendez vous et défendre ses ambitions pour la protection de ce bien commun, comme le souligneront les dirigeants européens à Bruxelles.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la violence de l’agression russe contre l’Ukraine, puis la fermeté, pour ne pas dire la brutalité, du président Trump, ont provoqué un véritable réveil européen. Secoués de la torpeur dans laquelle nous avaient plongés les dividendes de la paix, nous n’avons pas d’autre choix que d’assumer notre propre sécurité. Comme l’a dit le président Perrin lors du débat que nous avons eu la semaine dernière au Sénat, il nous revient maintenant de « diffuser en Europe notre volonté d’indépendance et de souveraineté ». Les conclusions du dernier Conseil européen extraordinaire vont dans le bon sens. L’Union européenne semble déterminée à accroître sa préparation globale en matière de défense et à combler ses lacunes. Elle semble aussi vouloir y mettre les moyens. Qu’y a t il toutefois, à ce stade, derrière les mots ? Le dernier Conseil européen a validé le paquet de mesures exceptionnelles proposées par la présidente de la Commission, qui visent à financer un surcroît de dépenses de défense estimé à 800 milliards d’euros. Le montant est impressionnant. Il correspond exactement aux 5 % du PIB des États membres exigés par le président Trump. D’aucuns feront sans doute remarquer que l’on s’autonomise en obéissant… Cependant, au fond, seul l’objectif compte, à condition toutefois que l’on se donne les moyens de l’atteindre. d’abord, d’être plus précis. Le ministre Barrot a dit que la France se saisira de tous les instruments que la Commission mettra sur la table, tels que la dérogation aux règles budgétaires, les facilités de prêt ou encore l’emploi des fonds de cohésion inutilisés. Nous aimerions toutefois avoir davantage de détails sur les montants en jeu et sur leur emploi. Ensuite, on ne voit pas encore bien comment garantir que cet effort de défense profitera prioritairement à l’industrie européenne. Le projet de règlement Edip, qui est en cours de discussion, ne représente encore qu’une goutte d’eau dans l’océan des investissements nécessaires et ne prend pas exactement le plus court chemin pour réduire nos dépendances à l’industrie américaine. La méthode retenue pose d’autres problèmes. La présidente de la Commission invoque, pour accélérer la mise en œuvre des nouveaux instruments, l’article 122 du traité sur le fonctionnement de l’Union

Une autre question reste lancinante : s’agit il d’un plan pour renforcer la défense européenne, ou bien d’un moyen d’accroître le contrôle, par les institutions européennes, de la défense des États européens ?

Une telle mesure appelait forcément à son tour une riposte américaine sur les vins et spiritueux européens. Celle ci, cette fois, expose bien davantage l’économie française.

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues,

pour les océans, visant à favoriser la résilience des océans face au changement climatique, à promouvoir une économie bleue compétitive et à développer la connaissance et la recherche relatives aux écosystèmes marins. Ce pacte pourrait également comporter des mesures législatives afin d’aider les communautés côtières et rurales dépendantes des océans à gérer les

Afin de préparer ce pacte, la Commission européenne a sollicité l’avis des parties intéressées en début d’année. La France, qui possède le deuxième domaine maritime au monde, se doit d’être aux avant postes des négociations européennes sur les politiques maritimes et littorales. ministre, comment envisagez vous le rôle de la France dans l’élaboration du pacte européen pour les océans, et quelles priorités allez vous mettre en avant ? La France bénéficie d’un espace maritime de près de 11 millions de kilomètres carrés, répartis entre quatre océans, et dont 97 % se situent en outre mer. Les territoires ultramarins sont donc stratégiques, et je dirais même incontournables, dans la protection et la mise en valeur du patrimoine marin de notre pays. Ils sont également en première ligne face aux phénomènes climatiques extrêmes, comme l’actualité récente l’a encore démontré de manière dramatique. Ils sont aussi très exposés à la criminalité en mer : la pêche illicite, la piraterie ou encore le narcotrafic. Monsieur le ministre, de quelle manière la France met elle en avant les enjeux et les besoins spécifiques des outre mer dans la conception du pacte européen pour les océans ? Quels instruments pourrions nous promouvoir pour permettre à ces territoires de jouer un rôle actif dans la mise en œuvre de ce futur outil ? J’en arrive à mon second point : alors que la haute mer représente plus de 60 % de la surface des océans

Cet accord historique a été signé par 111 États depuis le mois de septembre 2023, ce qui traduit, je m’en réjouis, une réelle volonté politique de la communauté internationale de poser les bases d’une conservation et d’une utilisation durables des écosystèmes marins,

qui prévoit la protection d’ici à 2030 d’au moins 30 % des mers et des océans. Pour que le traité entre en vigueur, il doit être ratifié par au moins soixante États signataires. C’est chose faite pour la France, grâce à l’adoption par le Parlement, à l’unanimité, du projet de loi autorisant cette ratification, en novembre 2024.

la première zone économique exclusive au monde, grâce notamment à ses régions ultrapériphériques. Ce pacte doit être ambitieux, aligné avec les autres cadres mondiaux et régionaux. Il doit servir de modèle en matière de préservation de l’océan, pour promouvoir une approche globale, comprenant les enjeux liés à la biodiversité,

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, alors que la menace ne faiblit pas sur le front ukrainien et que l’allié américain vacille, il appartient à l’Union européenne d’être ferme, de s’opposer à l’agression russe et de permettre à ses États membres d’assurer la sécurité sur le continent. En tant que rapporteur général de la commission des finances du Sénat, ma responsabilité est aussi de veiller à ce que cet effort soit soutenable pour la France. La prochaine réunion du Conseil européen permettra d’avancer sur ce point et de préciser les annonces qui se sont succédé ces dernières semaines sur la constitution et le financement d’une Europe de la défense.

La Commission européenne a d’abord fait part de son intention d’activer la clause de sauvegarde prévue dans le pacte de stabilité et de croissance. Cela lui permettrait d’exclure, dans son calcul du déficit public, les dépenses engagées par les États membres en matière de défense, jusqu’à 1,5 % de leur PIB. Si je salue la latitude accordée par les institutions européennes aux États membres, afin d’apporter une réponse à la hauteur des enjeux, je me dois de rappeler ici une évidence : une telle disposition ne desserre en rien la contrainte financière qui pèse sur notre pays.

et les Français, et cela demeurera. Monsieur le ministre, comment comptez vous concilier une hausse de notre effort militaire avec la nécessaire maîtrise du déficit et de la dette de notre pays ? J’en viens à la seconde proposition forte de la Commission européenne, à savoir un nouvel instrument visant à accorder 150 milliards d’euros de prêts aux États membres pour des investissements dans le domaine de la défense. dernières informations, les emprunts se feraient sur une base volontaire et nécessiteraient que les États se mettent au moins à deux pour investir dans les domaines où les besoins sont les plus urgents : défense aérienne, drones, artillerie, munitions, etc. Pouvez vous m’indiquer la position que vous défendrez dans la définition des contours de ce nouvel instrument ? Si ces emprunts sont bien accordés sur une base volontaire et dans les conditions que je viens d’exposer, la France souhaite t elle recourir à ce dispositif et, si oui, à quelle hauteur et pour quelles dépenses ? Si les contours de cet instrument doivent être discutés lors du prochain Conseil, il apparaît à ce stade non pas comme un nouvel emprunt commun au niveau de l’Union européenne, sur le modèle de ce qui avait été fait pour le plan de relance, mais plus comme une façon pour les États membres de lever une dette supplémentaire en passant par la Commission européenne. Quel est l’intérêt d’un tel dispositif pour la France ?

Cette réunion est importante, puisqu’elle permettra aux chefs d’État et de gouvernement d’évoquer les initiatives que la Commission européenne commence à déployer au travers de certaines communications stratégiques, comme la boussole de compétitivité, ou de paquets de simplification dits omnibus. Ces orientations visant à simplifier, à alléger le fardeau réglementaire, à mieux prendre en compte les réalités économiques et les besoins des territoires sont une nécessité, comme le Sénat l’a souligné à de nombreuses reprises. Je pense notamment à la prise en compte des réalités des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire,

esquissée par la Commission européenne et je veux saluer les premières annonces de simplification qu’elle a faites en matière de durabilité ou de mécanisme d’ajustement carbone

Nous irons défendre nos positions à Bruxelles pour que la Commission fasse preuve de plus d’audace, le contexte international dans lequel nous évoluons ayant fondamentalement changé. Les rapports des anciens premiers ministres italiens, Enrico Letta et Mario Draghi, que vous avez rappelés, monsieur le ministre, ont souligné les défis à relever. nous avons pu mesurer, lors d’une récente conférence interparlementaire à Bruxelles, que faire bouger les lignes n’allait pas de soi et que les paroles étaient diverses au sein des États membres. Ce Conseil européen apparaît aussi comme une réunion de transition, de transition, d’abord sur la question du financement de l’industrie de défense, après la réunion extraordinaire du Conseil européen du 6 mars. À mes yeux, la réponse ne pourra pas seulement provenir des fonds publics : nous devons pousser les feux sur la mise en place de l’Union pour l’épargne et l’investissement, mais aussi faire en sorte que la Banque européenne d’investissement joue un réel rôle de soutien du secteur de la défense. Nous en avons parlé ensemble la semaine dernière, Je crains par ailleurs que notre pays, compte tenu de sa situation budgétaire, ne soit pas en mesure de bénéficier massivement des assouplissements envisagés du pacte de stabilité et de croissance. Je m’interroge également, comme comme le rapporteur général Jean François Husson, sur l’intérêt qu’il pourrait trouver à solliciter l’enveloppe de prêts envisagée par la Commission, à hauteur de 150 milliards d’euros. Cette réunion est également une réunion de transition dans le cadre de la préparation du prochain cadre financier pluriannuel. L’Union européenne fait face à des besoins croissants et nous refusons de remettre en cause les politiques traditionnelles, comme la politique de cohésion et la politique agricole commune. Aucune porte de sortie n’ayant pour l’instant été trouvée dans le dossier des ressources propres, l’équation actuelle est intenable et il faut trouver une solution. La présidente de la Commission européenne déclarait la semaine dernière que le temps des illusions était révolu. Il est temps, en effet, de repenser réellement un certain nombre de politiques européennes, sans toutefois que cela soit synonyme de dessaisissement des États membres, Pascal Allizard. Pour le dire clairement, la Commission européenne doit agir avec plus de fermeté dans des domaines où elle est réellement compétente. Je pense à la réponse à la hausse des tarifs douaniers décidée par le président des États Unis, à la lutte contre la concurrence déloyale dans les relations commerciales ou à la mise en œuvre des règlements européens, que les grandes plateformes du numérique doivent respecter. Monsieur le ministre, pouvez vous nous confirmer que la France adoptera une ligne de fermeté sur ces sujets ? Très bien

le financement de nos entreprises : faisons en sorte que le marché unique soit véritablement une opportunité pour nos PME, nos entrepreneurs, nos innovateurs. À cet

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le Conseil européen qui se tiendra les 20 et 21 mars prochain revêt une importance toute particulière. En quelques semaines, le président des États Unis et ses acolytes ont, hélas ! plongé le monde dans une instabilité dangereuse. Il y a eu la séquence ahurissante du 28 février dernier, au cours de laquelle nous avons été témoins de l’humiliation infligée par Donald Trump à Volodymyr Zelensky, suivie du lâchage en pleine guerre des Ukrainiens, le tout assorti d’un narratif scandaleux et de leçons de morale données par J.D. Vance aux Européens à Munich sur la liberté d’expression. Je n’oublie pas les déclarations tonitruantes sur l’annexion du Groenland et du Canada. Faut il être surpris de voir l’homme de la Maison Blanche aujourd’hui brutaliser ses concitoyens au mépris de la Constitution, désarmer tous les contre pouvoirs, laisser son double maléfique, Elon Musk, s’attaquer au démantèlement de l’État et des agences fédérales, tout en se mêlant de nos affaires ? En trahissant ou agressant les traditionnels alliés des États Unis, en s’alignant sur le Kremlin, Donald Trump a fait voler en éclats l’ordre issu de la Seconde Guerre mondiale. Comme si cela ne suffisait pas, il est par ailleurs en train de plonger les échanges et les paiements mondiaux dans le chaos, tout en déstabilisant l’économie américaine qui, pourtant, se portait plutôt bien. La collusion du pouvoir avec les illuminés de la tech, qui font désormais la loi, accentue encore un peu plus ce que nous avons maintes fois dénoncé ici : ce capitalisme de prédation et de surveillance, hors de toute règle et de toute éthique, qui a poussé l’Union européenne à poser des règles pour son propre territoire. L’Europe est donc aujourd’hui renvoyée à elle même, prise en tenaille entre la Russie, la Chine et les États Unis. Désormais, c’est le sursis ou le sursaut ! Il n’y a pas d’autre choix que de se réarmer militairement, mais aussi politiquement et économiquement. Notre ministre des armées dit juste : pour commencer à se réarmer, il faut que chacun des États membres trouve les voies et moyens de faire les efforts qui s’imposent, tout en pensant une nouvelle architecture de sécurité comprenant, bien évidemment, le Royaume Uni qui, comme la France, dispose de la dissuasion nucléaire. Dans ce contexte, je salue l’annonce d’Ursula von der du lancement du programme ReArm Europe, qui pourrait mobiliser près de 800 milliards d’euros. En attendant, l’urgence, c’est de collectivement soutenir l’Ukraine avec nos alliés. À ce jour, l’Union européenne lui a fourni 135,4 milliards d’euros, dont 49,2 milliards de soutien militaire, de subventions, d’aides en nature et de prêts à des conditions très favorables. En 2025, elle fournira 30,6 milliards d’euros au titre de la facilité pour l’Ukraine et au titre du prêt extraordinaire accordé par le G7 et financé par les avoirs russes alors que Donald Trump et Vladimir Poutine continuent à discuter d’une possible trêve, la France doit réaffirmer que toute trêve ou tout cessez le feu ne peut avoir lieu que dans le cadre d’un processus menant à un accord de paix global. Il ne peut y avoir de négociations affectant la sécurité européenne sans la participation de l’Europe. Il ne peut y avoir de négociations sur l’Ukraine sans l’Ukraine. Celle ci ne saurait d’ailleurs payer au prix fort une guerre qu’elle n’a pas déclenchée. L’Europe devra surtout s’assurer que les accords de paix soient respectés pour ne pas subir un nouveau conflit à court terme. Souvenons nous des accords de Minsk en 2014 ! Il faut des garanties de sécurité robustes et crédibles pour l’Ukraine, et au delà pour nous mêmes, car, ne nous leurrons pas, le plan de Poutine est de revenir au partage du monde décidé à Yalta. Selon les évaluations de l’Otan, de l’Allemagne, de la Pologne, du Danemark et des États baltes, la Russie pourrait être prête à attaquer un pays de l’Union européenne d’ici trois à dix ans. Alors, il s’agit bien de dissuader Poutine de revenir à la charge. Pour cela, l’Union doit aussi se réarmer politiquement. Pour être efficace, compétitive et répondre aux défis du moment, elle doit être plus politique que bureaucratique, plus stratège que tatillonne. À cet égard, je vous renvoie, monsieur le ministre, au rapport que nous avons réalisé avec le président Rapin sur la dérive normative de l’Union, également pointée du doigt

Personnellement, j’alerte depuis plus de dix ans sur l’urgence à construire autre chose qu’une simple Europe des consommateurs : une Europe des acteurs. Qu’on le veuille ou non, l’internet est un terrain d’affrontement mondial pour la domination du monde par l’économie et la connaissance. Théâtre de cyberattaques en tout genre, toujours plus nombreuses, c’est un terreau fertile pour la guerre informationnelle et les ingérences étrangères. Si ses chars ne sont pas aux portes de Paris, la Russie nous livre bien une guerre cyber souterraine. L’Union a enfin légiféré utilement ces dernières années pour protéger les données des Européens, un actif stratégique majeur, pour créer les conditions d’un marché plus équitable pour nos propres entreprises face à la concurrence des, pour réguler les services proposés par ces plateformes au modèle toxique, pour soutenir le développement d’une intelligence artificielle de confiance, mais elle a failli industriellement, empêchant ainsi toute souveraineté numérique. Alors, monsieur le ministre, je reprends la formule de l’un de mes nombreux rapports : il est plus que temps de reprendre en main notre destin numérique ! Nous venons d’adopter le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, transposition de la directive NIS 2, qui établit une véritable architecture de sécurité pour notre pays, nos entreprises, nos collectivités territoriales et entités critiques. C’est très bien d’appliquer certains standards, encore faut il le faire en ayant recours à des entreprises françaises et européennes imperméables aux lois extraterritoriales américaines ou chinoises et dont nous serons sûrs. Rehausser notre sécurité en ligne, c’est aussi du réarmement : à ce titre, les dépenses effectuées devraient pouvoir échapper aux règles du pacte de stabilité et de croissance. Le marché va se développer : il faut en profiter pour soutenir notre filière cyber, notamment par le levier de la commande publique avec la réforme annoncée de la directive sur les marchés publics en 2026. C’est bien ce qu’ont su faire les Américains, les Russes et les Chinois. Ma collègue Florence Blatrix Contat et moi même l’avons encore martelé ces derniers jours en proposant au vote de la commission des affaires européennes plusieurs propositions. Nous avons notamment appelé à la création d’outils souverains fondés sur des règles éthiques rigoureuses et sur le mode qui soient de véritables substituts aux modèles toxiques des plateformes, ainsi qu’à un investissement massif dans les dernières technologies, l’intelligence artificielle et le quantique, dans le cadre du programme Horizon Europe. Nous demandons aussi la stricte et rigoureuse application des règlements européens portant sur la régulation du numérique, n’en déplaise à MM. Musk et Zuckerberg, dont le combat au nom de la prétendue liberté d’expression justifie le non respect de la loi et toutes les dérives sur les réseaux sociaux, y compris les plus graves : celles qui mettent en danger nos enfants, conduisent à l’assassinat d’un professeur, ou encore menacent nos démocraties au travers de la manipulation des opinions et des élections. Il faut à cet égard que le bouclier européen de la démocratie annoncé par la Commission européenne soit adopté rapidement. Il devra renforcer les moyens de contrôle des plateformes numériques, en particulier en fixant des normes éthiques minimales tous les algorithmes de recommandation, et ce dès leur conception. Il faut aussi qu’il garantisse la pérennité et la vitalité de nos médias et du journalisme

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l’heure où l’Europe s’apprête à se réunir pour un Conseil déterminant, une certitude s’impose : l’avenir du continent se joue sous nos yeux.

Si nous approuvons la nécessité de soutenir le peuple ukrainien, victime d’une guerre atroce et injustifiable choisie par Vladimir Poutine, nous affirmons aussi que la paix ne se construit pas dans l’escalade. Pourtant, c’est bien cette voie qui est choisie, avec une nouvelle annonce du ministre des armées évoquant un « poids de forme » de l’armée à 90 milliards d’euros, contre 50 milliards aujourd’hui, un triplement annoncé des dépenses militaires européennes, des prêts garantis par l’Union européenne à hauteur de 180 milliards d’euros et une obsession martiale qui fait écho aux mots glaçants de Mme von der Leyen : « Le temps est venu d’assurer la paix par la force. Nous soulignons le paradoxe suivant : à l’heure où la paix se construit difficilement dans une ébauche de cessez le feu, l’Union appelle au surarmement, avec 800 milliards d’euros mobilisés sur plusieurs années, soit 5 % du PIB européen. Ce chiffre résonne étrangement avec les exigences de Donald Trump, qui veut voir l’Otan financée par l’Europe, tout en conservant la suprématie américaine. Mme von der Leyen lui offre finalement sur un plateau ce qu’il réclamait depuis des années. Autre coïncidence, c’est aussi le montant avancé par Mario Draghi pour sauver la compétitivité européenne. Vous ne pourrez pas cacher éternellement cette réalité : l’Europe est aux armes américaines. Les importations d’armes par les pays européens membres de l’Otan ont plus que doublé entre les périodes 2015 2019 et 2020 2024. Dans le même temps, les États Unis nous ont fourni 64 % de ces armes, contre 52 % auparavant. En clair, nous importons deux fois plus d’armes et nous sommes toujours plus dépendants des États Unis. Monsieur le ministre, dans l’attente d’une Union pour l’épargne et l’investissement, devrons nous compter sur BlackRock et consorts pour accompagner la base industrielle et technologique de défense française ? défense française ? Nous ne croyons pas en cette doctrine qui transforme l’Europe en machine de guerre. Nous ne croyons pas à cette fuite en avant, où les dividendes des marchands d’armes explosent pendant que l’on demande aux peuples de se serrer la ceinture.

La France ne doit pas être l’otage de cette stratégie de militarisation à marche forcée. Il est temps d’engager une autre voie, celle d’une conférence d’Helsinki 2 imaginant une nouvelle sécurité collective qui ferait de l’Europe non pas un terrain de manœuvres militaires, mais un pôle de stabilisation et de diplomatie. La question ukrainienne ne peut évidemment occulter les grandes tensions qui traversent le monde, à commencer par le Proche Orient et le Moyen Orient. La situation en Syrie, avec le massacre de plus d’un millier de civils alaouites, mais aussi de chrétiens, ne laisse pas de nous interroger sur la fiabilité des nouvelles autorités de ce pays et sur la crédibilité de la conversion à la démocratie de leurs dirigeants. C’est bien sûr la situation en Palestine, à commencer par Gaza, qui continue à nous préoccuper au plus haut point. Les trêves se suivent, sans lendemain, et le sort des derniers otages, ou de leurs cadavres, n’est toujours pas réglé. La responsabilité porte à la fois sur le gouvernement Netanyahou, allié à l’extrême droite, et sur l’islamisme radical, qui pollue la juste cause palestinienne. Comment la diplomatie européenne peut elle, dans cette situation inextricable, agir de façon efficace, si ce n’est, comme l’a déjà fait l’Espagne, en reconnaissant deux États, Israël et la Palestine ? Enfin, je veux conclure sur ceux qui, chez nous, subissent les logiques d’intérêts à courte vue de l’Union européenne. Les salariés du Pas de Calais, des Hauts de France et d’ailleurs savent ce que veut dire dire le mot « compétitivité ». Ce fut l’argument pour briser les mines, le textile, la sidérurgie. Aujourd’hui encore, c’est l’excuse parfaite pour justifier la fermeture d’usines, les suppressions de postes, la disparition des savoir faire et l’allégement du devoir de vigilance, comme le prévoit d’ailleurs la nouvelle directive omnibus. La parole

L’Union européenne nous a permis de créer un continent de paix, de coopération, remplaçant des siècles de violences, de conflits, de nationalismes par le dialogue, le droit et la régulation, mais nous avons toujours des voisins

Les illusions se dissipent et chacun voit bien que c’est le principe même de l’Union européenne qui est attaqué au travers de l’agression et des prétentions russes contre la liberté du peuple ukrainien. Avec cette montée du recours à la force et à la violence comme méthode principale d’acteurs étatiques et non étatiques, c’est notre modèle européen fondé sur la coopération, la régulation et le droit, modèle porteur de nos valeurs de démocratie et de liberté, qui est attaqué. Voilà ce à quoi les États Unis d’Amérique et leur Président erratique et autoritaire sont dorénavant hostiles ! L’Europe est au pied du mur, condamnée à l’impuissance, voire à la dislocation, si elle n’accomplit pas l’indispensable saut fédéral seul à même d’assurer sa sécurité collective et celle de l’Ukraine en première ligne, si elle n’engendre pas cette Europe de la défense – défense de ses valeurs, défense de ses intérêts. L’écologie politique porte le pacifisme au cœur de son histoire. Nous ressentons donc l’anxiété populaire face à cet engrenage militaire, mais nous affirmons d’autant plus nettement qu’il nous faut admettre le rapport de force pour préserver notre sécurité et nos idéaux, pour préserver l’espérance du droit international et du multilatéralisme. Les fortes paroles et les résolutions prises nécessitent que des actes soient engagés. C’est ce que nous attendons de ce Conseil européen. Il ne peut être question de « limiter notre niveau de préparation à ce qui est aisé à obtenir politiquement » ; il convient de répondre aux besoins pour faire face aux scénarios les plus graves. Si la Hongrie ou la Slovaquie s’obstinent à se désolidariser de l’aide à l’Ukraine l’Ukraine et à contrecarrer la construction de l’Europe de la défense, il faudra bien que les autres États membres fassent progresser le vote à la majorité qualifiée, au lieu de l’unanimité aujourd’hui requise dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité. et de sécurité. Pour répondre aux défis du temps présent, il nous faut sans doute remettre en cause le cadre de gouvernance qui limite les ressources financières : il s’agit de garantir une sécurité de financement à long terme

les bénéfices exceptionnels des acteurs systémiques du secteur de la défense. Pour financer le plan de 800 milliards d’euros annoncé, il faudra avant tout créer de nouvelles ressources propres plutôt que de chercher ces sommes dans les fonds de cohésion ou dans ceux de la politique agricole. Il serait désastreux de s’aliéner nombre de citoyens européens en mettant en concurrence les investissements dans la défense avec les dépenses sociales, la cohésion territoriale et la transition climatique. Seul le renforcement du tissu social et économique de l’Europe renforcera la capacité de l’Union à se défendre contre la désinformation et l’influence étrangère. Ne donnons pas davantage de grain à moudre au réseau X, aux médias Bolloré, ou encore à des forces politiques fascinées par Poutine ou par Trump ! Bâtir notre autonomie stratégique n’est pas seulement une question d’armes et de munitions. Il importe de sortir de cette logique contre productive qui a fait que, en 2024, alors que nous donnions d’une main 19 milliards d’euros à l’Ukraine, nous en versions de l’autre 22 milliards à la Russie en échange de ses énergies fossiles ! La transition énergétique et le Pacte

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, à l’approche du Conseil européen des 20 et 21 mars, ce débat préalable devant la représentation nationale est d’autant plus essentiel que l’actualité internationale ne cesse de se dégrader. Les défis majeurs qui attendent l’Europe comme l’a déjà montré le Conseil européen extraordinaire présidé par Antonio Costa le 6 mars dernier. Au cœur des débats européens figurent évidemment la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et la question de la défense européenne, mais aussi la politique migratoire et, plus largement, notre politique extérieure. Malgré la poursuite des pressions russes et une position américaine instable, tournée d’abord vers ses propres intérêts, l’Ukraine continue de se battre vaillamment pour sa souveraineté. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain tient à réaffirmer ici son plein soutien à la résistance ukrainienne et à sa mobilisation pour une paix juste et durable. Les sénateurs et députés socialistes restent favorables à la saisie sans délai des 210 milliards d’euros d’avoirs russes gelés et immobilisés, ainsi qu’à l’affectation intégrale à l’Ukraine des intérêts qu’ils produisent. C’est aussi la position adoptée par la majorité de l’Assemblée nationale. Laisser fléchir notre engagement aux côtés de l’Ukraine serait non seulement trahir un peuple agressé, mais aussi exposer toute l’Europe à de nouvelles menaces, physiques et cyber. Alors, monsieur le ministre, le Gouvernement compte compte t il, enfin, porter cette exigence de justice devant le prochain Conseil européen et soutenir plus fermement la confiscation des avoirs russes et leur réaffectation directe au renforcement militaire de la résistance et à la reconstruction de l’Ukraine ? Nous observons évidemment les différents mouvements du Président de la République et les efforts qu’il a déployés conjointement avec le Premier ministre britannique. Mais pouvez vous nous assurer que, au delà de cette implication toute personnelle d’Emmanuel Macron,

Alors que le Brexit a malheureusement modifié la place des Britanniques dans l’Europe, pouvez vous nous indiquer quelles seront les prochaines étapes du rétablissement de relations franco allemandes plus fidèles à l’histoire de la construction européenne ? Face aux États plus frileux, le moteur franco allemand nous paraît en effet stratégique pour renforcer, d’urgence, l’action politique, économique et militaire de l’Europe. Celle ci doit se placer en première ligne face aux conflits qui secouent le monde et aux menaces qui pèsent sur la paix globale. Quant à la France, elle doit peser de tout son poids pour que l’Europe se crée une place, non pas contre les États Unis ou quiconque d’autre, mais pour elle même, pour sa sécurité et notre avenir à tous. C’est vrai des négociations d’une trêve éventuelle entre l’Ukraine et la Russie. C’est vrai face à la situation sensible dans les Balkans. C’est vrai aussi des prochaines étapes du cessez le feu au Proche Orient. Les négociations entre Israël et le Hamas semblent piétiner et les États Unis s’imposent dans la région y jouer un rôle dont chacun perçoit bien la dangerosité et la faible compatibilité avec nos valeurs. Dans ce contexte, pouvez vous nous dire, monsieur le ministre, quelle initiative précise la France entend prendre, en lien avec l’Union européenne, pour exercer une influence positive en faveur d’une résolution juste et rapide de ce conflit meurtrier

Au regard de l’obsession migratoire de votre collègue ministre de l’intérieur Bruno Retailleau, il faut reconnaître, monsieur le ministre, que nous ne sommes malheureusement guère surpris du silence de la France sur les aspects les plus préoccupants de ce projet de règlement, qui comporterait de graves atteintes au droit d’asile et au principe de non refoulement Allez vous réellement laisser faire, ou pouvons nous compter sur votre discernement pour que la France veille à ce que ce nouveau texte, préparé à la hâte, sans concertation réelle avec les ONG,

L’Europe ne peut pas, d’un côté, prôner le respect des droits humains partout dans le monde et, de l’autre, accepter les « de retour » et accréditer la thèse selon laquelle les migrants seraient d’abord des criminels devant être traités comme tels.

par ces actifs, les profits d’aubaine, sont aujourd’hui utilisés pour financer un prêt de 50 milliards d’euros du G7 à l’Ukraine, qui sert à financer à la fois ses besoins macroéconomiques et ses besoins militaires. L’Union européenne couvre 20 milliards d’euros de ce prêt

d’une relance du dialogue politique qui pourra mener à deux États, israélien et palestinien, à la sécurité des Israéliens, à la souveraineté des Palestiniens et à la libération sans condition de tous les otages. La diplomatie française a été particulièrement mobilisée sur ce dossier. Elle a également joué, aux

une guerre se déroule sur notre continent ; notre principal allié semble n’en être plus un ; notre économie est fragilisée. C’est dans ce contexte que se tiendra la réunion du Conseil européen

un million de personnes massacrées, mutilées, sacrifiées sur l’autel de l’impérialisme russe. Alors que les États Unis de Donald Trump ont fait le choix de se rapprocher de celui qui a provoqué cette guerre, l’Europe doit, plus que jamais, être mobilisée. Le 6 mars dernier, le Conseil européen s’était réuni pour une session extraordinaire à la suite de la suspension de l’aide américaine à l’Ukraine. À cette occasion, les Vingt Sept se sont accordés sur des mesures historiques pour la défense européenne. Cependant, de nombreux points restent en suspens. Sur l’Ukraine, la position commune adoptée le 6 mars renvoie à la « prochaine réunion » du Conseil européen. En effet, la Hongrie de Victor Orban, soutien de Donald Trump, a refusé d’approuver les positions des vingt six autres États membres en faveur du renforcement du soutien du soutien à l’Ukraine. Le groupe Les Indépendants le déplore et fait part de ses vives inquiétudes sur l’attitude de la Hongrie. Monsieur le ministre, pourriez vous nous faire un point d’étape sur ce sujet déterminant pour notre sécurité collective et nos valeurs ? En Syrie, l’histoire semble se répéter. Les tensions communautaires, qui déchirent le Proche Orient depuis des décennies, ont encore donné lieu à des violences d’une brutalité inouïe. En l’espace de quatre jours, des milliers de civils ont été assassinés et blessés. Des forces armées islamistes, liées au groupe Hayat ont massacré des populations chrétiennes et alaouites, la communauté du dictateur Bachar al Assad. Ces assassinats de masse rappellent les représailles dont ont fait l’objet les sunnites après la chute de Saddam Hussein, puis les chiites lors de l’arrivée de Daech. Ils font craindre le pire pour la Syrie. Quelle est la réponse de l’Union européenne face à cela ? Aujourd’hui même, l’Union organise à Bruxelles la neuvième conférence à la Syrie, afin de lever des fonds pour soutenir le peuple syrien. Il y a moins d’un mois, elle avait décidé de suspendre un certain nombre de sanctions prises à l’encontre de la Syrie, tout en réaffirmant sa volonté d’être aux côtés du peuple syrien dans la période de transition qui s’ouvre pour lui. La Syrie a réussi à se libérer du joug de Bachar al Assad, mais le combat n’est pas terminé. Aujourd’hui, des Syriens risquent leur vie en raison de leur appartenance religieuse ; je pense notamment aux chrétiens d’Orient. Ne laissons pas se reproduire ce qu’il s’est passé en Irak ! La situation appelle une vigilance absolue, et l’Europe devra être au rendez vous. Au delà de la guerre, c’est notre économie qui est aujourd’hui menacée. Paru en septembre dernier, après celui de M. Letta, le rapport de M. Draghi sur notre compétitivité est sans appel. Pour qualifier la situation de l’économie européenne, Mario Draghi en vient à parler de « lente agonie ». Or qui dit affaiblissement économique dit perte de souveraineté et d’indépendance. C’est pourquoi la compétitivité européenne sera, elle aussi, au cœur des échanges des 20 et 21 mars. La Commission européenne semble

Le groupe Les Indépendants salue cette démarche, mais insiste sur la nécessité de prioriser les initiatives visant à simplifier les normes. Cette simplification est vitale pour l’avenir de nos entreprises. Elle est d’ailleurs au cœur des priorités de l’Union, comme le de l’Union, comme le montre le paquet législatif omnibus dévoilé à la fin du mois de février. Dans un monde de plus en plus instable, face à une concurrence de plus en plus déloyale, ces mesures de simplification s’imposent. Il y va de notre souveraineté. En ce sens, monsieur le ministre, comment envisagez vous la mise en œuvre de ces mesures à l’échelle nationale ? Les 20 et 21 mars, le Conseil européen abordera également le prochain cadre financier pluriannuel Cette question est tout aussi stratégique pour notre souveraineté que la compétitivité. Le 12 février dernier, la Commission a présenté un document exposant les grandes orientations de ce prochain budget. Pour sa part, le groupe Les Indépendants alerte sur la nécessité d’un budget qui soit à la hauteur des défis qu’il nous faudra

irrégulière. En effet, chaque année, près d’un demi million de migrants illégaux reçoivent l’ordre de quitter l’UE, mais seulement un sur cinq le fait. Comment faire respecter notre politique migratoire si notre droit n’est pas réellement appliqué ? Nous accueillons donc cette volonté de réforme. Dans ce domaine, monsieur le ministre, quelles sont les perspectives du Gouvernement ? Pour conclure, j’insiste sur le moment de bascule historique dans lequel nous nous trouvons. Notre seule boussole doit être le renforcement, l’unité et l’efficacité de l’Union européenne. C’est ce que notre groupe attend de la prochaine réunion du Conseil

Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, en l’espace de trois ans, l’environnement stratégique du continent européen s’est radicalement transformé. D’abord, c’est un tabou que la Russie a brisé, en recourant à la force armée contre un État voisin et en violant ses frontières pour les remodeler. Désormais, c’est le totem de l’alliance atlantique que le Président américain fait vaciller au travers de son rapprochement avec Vladimir Poutine, de ses critiques envers l’Otan, de ses attaques sur le terrain commercial. Pour nombre de pays européens qui ont assis leur vision du monde, leur prospérité et leur sécurité sur le lien transatlantique, l’émotion est particulièrement vive. Pourtant, la situation exige avant tout une analyse lucide, que ce soit sur l’état de la menace ou sur celui de nos alliances. En effet, alors que l’armée russe jette toutes ses forces dans la bataille et que ses pertes humaines et matérielles atteignent des niveaux considérables, ses avancées restent modestes. Et si, après trois ans de combats, elle n’a pas réussi à passer le Dniepr, qui pourrait croire qu’elle est en mesure de se porter jusqu’aux rives du Rhin ? Néanmoins, le passé récent, en Géorgie ou en Ukraine, alimente les craintes de nos amis et alliés d’Europe centrale. Par ailleurs, nous ne pouvons ignorer les risques que la Russie fait peser sur notre pays, que ce soit par ses intimidations nucléaires et balistiques ou par l’agressivité qu’elle manifeste à notre encontre dans tous les champs hybrides. La menace russe est donc objective. La qualifier d’existentielle, comme l’a fait le Président de la République, est à mon sens tout à fait exagéré, mais il n’en reste pas moins vrai qu’elle s’est renforcée et qu’elle trouve dans le nouveau positionnement américain un contexte favorable à son intensification. Quant aux États Unis, ils sont certes devenus un allié imprévisible, mais ils restent tout de même un allié. Ainsi, ni une dénonciation de l’article 5 du traité de l’Atlantique Nord ni un retrait des dizaines de milliers de soldats américains stationnés en Europe ne semblent devoir advenir dans un avenir proche. pas moins : le pivot des États Unis vers l’Asie s’accélère. Et demain, indépendamment de la présidence Trump, l’engagement américain sur notre continent ne sera plus celui d’hier. Les Européens sont dès lors face à un choix. Il ne s’agit pas de penser notre sécurité collective en dehors de toute alliance ni, encore moins, de se préparer à affronter la Russie sur le terrain ukrainien. Aucune de ces extrémités n’est raisonnable ni même crédible. Il importe en revanche de prendre acte des transformations de l’ordre international et des bouleversements de notre environnement proche, et d’agir en conséquence, ne serait ce que pour gagner la considération stratégique qui nous est aujourd’hui refusée. À court terme, cela signifie que nous ne pouvons abandonner l’Ukraine à son sort. À moyen et long terme, cela impose de mettre enfin sur pied une défense du continent européen qui, pour être dissuasive, devra être à la fois crédible et autonome. Ne nous payons toutefois pas de mots : les défis à relever pour atteindre ces objectifs sont immenses. Cela prendra nécessairement plus de temps que nous ne le souhaiterions. Surtout, ils impliqueront d’agir selon certains principes. Je pense tout d’abord au pilotage de nos efforts collectifs. En effet, la remontée en puissance de nos outils militaires ne peut être menée anarchiquement ; elle devra nécessairement être coordonnée dans de nombreux domaines. Néanmoins, ce processus ne peut servir de paravent à la transformation des compétences dévolues par les traités. L’article 4 du traité sur l’Union européenne est parfaitement clair clair : « La sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre. » L’idée d’une armée européenne, à laquelle, heureusement, plus grand monde ne croit, est donc vouée à rester une chimère. Mais, au delà, nous devons affirmer que la coopération européenne de défense est par essence intergouvernementale et qu’elle doit le rester. Il n’est ainsi pas acceptable que la Commission européenne cherche, comme elle l’a fait dans le cadre de la proposition de règlement à s’arroger des prérogatives qui, par nature, ne peuvent pas être les siennes. De la sorte, la présidente von der Leyen dépasse à mon sens très largement ses attributions. En outre, les débats sur ce projet de règlement livrent un autre enseignement : la révolution culturelle qu’implique l’autonomie stratégique européenne n’est pas encore parvenue à son terme. En effet, si une certaine prise de conscience s’est indéniablement enclenchée, les discussions sur la notion de préférence européenne en matière d’achat de matériels militaires restent particulièrement difficiles, difficiles, en écho au fait que le réarmement qui a commencé à s’opérer en urgence dans les États membres s’est surtout concrétisé par des achats d’équipements américains. Or il y a là une contradiction majeure. Comment les Européens peuvent ils déclarer leur volonté d’assumer leur propre sécurité, voire proclamer leur souveraineté collective, tout en acceptant de rester sous tutelle, en étant armés par un tiers ? En ce qui nous concerne, la ligne est claire affirmer l’autonomie stratégique, c’est affirmer que la défense de l’Europe doit être assurée en premier lieu par les armes de l’Europe et que les fonds européens doivent aller aux entreprises européennes. Enfin j’évoquerai la dimension financière de ces enjeux. En effet, si nos efforts doivent s’amplifier, ils doivent aussi être financés.

En effet, loin de mettre sur la table 800 milliards d’euros d’argent frais, comme la présidente de la Commission aime à le faire penser, ce plan repose principalement sur deux propositions. D’abord, on exclurait, partiellement, les dépenses de défense des règles du pacte de stabilité et de croissance. Cette mesure, que nous soutenons de longue date, arrive bien tard, hélas ! car le déficit de la France atteint aujourd’hui des sommets, et s’il ne passe pas sous les fourches caudines de la Commission, il passera nécessairement tôt ou tard sous celles des marchés. Ensuite, le plan prévoit d’octroyer aux États membres des prêts garantis par le budget européen. Mais ceux ci devront bien être remboursés, tout comme d’éventuels nouveaux qui, en l’absence de nouvelles ressources propres, devraient être financés par les budgets nationaux. Pas plus pour la défense que pour d’autres secteurs, il n’y aura d’argent magique, et notre effort de défense ne pourra être assumé, pour l’essentiel, que grâce à des économies supplémentaires et à des réformes libérant le potentiel de croissance. Je me félicite ainsi que la Commission ait fait de la réduction de la charge administrative l’un des éléments clés de sa politique économique pour les cinq années à venir. Après des années passées à surréglementer méthodiquement, elle semble enfin avoir compris que la coupe était pleine pour nos entreprises, asphyxiées sous une avalanche de normes. Et nos industries de défense ne font pas exception, tant s’en faut. Il est donc positif qu’un train de mesures de simplification spécifiques à ce secteur accompagne la présentation cette semaine du livre blanc de la Commission. J’insiste néanmoins sur la nécessité absolue de revenir sur la conception de certains textes. Je pense en particulier à la taxonomie européenne des investissements durables, qui vient brider les circuits d’investissements et qui, il faut bien le dire, ressemble parfois à une mise à l’index pure et simple des entreprises de défense. Monsieur le ministre, mes chers collègues, le renforcement national et européen de nos outils militaires est une nécessité que nous reconnaissons sans ambages. Mais loin de l’émotion qui parfois peut nous saisir face au tourbillon des événements, cette tâche considérable exigera que nous nous y attelions avec calme et lucidité, avec détermination et constance – et surtout, monsieur le ministre, avec

renforcer la position de négociation des Ukrainiens dans le rapport de force avec la Russie, tout en réalisant des investissements massifs pour relancer notre outil de défense européen.

mes chers collègues, mercredi dernier, les ministres de la défense des cinq plus grandes nations militaires européennes – la France, l’Allemagne, la Grande Bretagne, l’Italie et la Pologne – étaient réunis à Paris. Nos objectifs sont toujours identiques faire front commun pour instaurer un nouveau cadre de sécurité pour l’Ukraine ; faire front commun avec une nouvelle politique de défense européenne ; faire front commun afin de répondre au rapprochement entre les États Unis et la Russie ; faire front commun au Parlement. Prenons le temps de nous rappeler les mots de celui qui, en 2017, entrait à l’Assemblée nationale et regardait avec mépris le drapeau européen présent dans l’hémicycle « On est obligés de supporter cela… », disait il ! Rappelons nous celle qui, en 2022, annonçait un recours devant le Conseil d’État parce que le drapeau européen flottait sous l’Arc de Triomphe, pendant la Présidence française du Conseil de l’Union européenne. C’était une provocation, à ses yeux ! Elle se disait défenseure des productions françaises, mais, dans le même temps, soutenait avec force celui qui envisage aujourd’hui d’imposer des droits de douane de 200 % sur le champagne et les vins français. Rappelons nous, au delà des symboles, qu’ils ont systématiquement été contre l’Europe et sa nécessaire souveraineté. Mais constatons aussi, dans le même temps, que le Président de la République a toujours poussé nos alliés à réfléchir à une défense commune et à investir

La volonté du chef de l’État a pu être critiquée, mais la politique s’inscrit dans le temps long, et l’ère géopolitique nouvelle qui s’est ouverte lui donne plus que jamais raison sur ce point. Certains aimeraient faire croire ici que nous aurions librement à choisir entre le réarmement et la défense de l’environnement, là que nous sommes en train de choisir le péril hypothétique russe plutôt que la lutte contre le terrorisme islamiste. Si nous comprenons aisément la raison politicienne et le ressort démagogique de ces discours, ils n’en restent pas moins faux et sont, en vérité, irresponsables. C’est bien parce que nous ne voulons, ni ne devons choisir que l’Europe unie est la solution, et la seule. Il en sera question lors du prochain Conseil européen, et il en sera question à titre principal – avec, bien entendu, la situation au Proche Orient. Dans ce contexte international bouleversé, grave, dangereux, anxiogène que nous connaissons désormais, nous avons ici même, au Sénat, débattu de la guerre en Ukraine à la veille de l’allocution présidentielle. si la défense nationale et les affaires internationales relèvent du domaine réservé du chef de l’État, le Parlement français jouera tout son rôle d’interpellation et de proposition, comme nous le faisons aujourd’hui. Monsieur le ministre, les dirigeants des Vingt Sept, soutenus par des majorités politiques très différentes, ont donné leur feu vert au plan de la Commission européenne pour nous réarmer contre les menaces expansionnistes et existentielles. La France a été motrice. Ce sont 800 milliards d’euros dont 150 milliards d’euros sous forme de prêts, pour renforcer nos capacités de défense. L’ancien ministre Hubert Védrine l’a souligné dans, c’est notre épreuve de vérité.

C’est pourquoi il a reçu les présidents de groupe de l’Assemblée nationale et du Sénat, au lendemain de l’adoption par les députés d’une résolution sur le renforcement du soutien à l’Ukraine. Mais il a démontré aussi,

que nous avons à débattre des projets de loi de programmation militaire, et que l’examen du prochain budget, sur ce point, sera d’une importance cruciale, pourriez vous nous détailler les positions que la France défendra ces 20 et 21 mars, sur le financement mutualisé et sur les outils prévus par chaque État membre ?

convoqué le 6 mars dernier, qui a surtout été l’occasion d’aborder la question du réarmement de l’Europe et de l’Ukraine dans le contexte géopolitique que l’on connaît. De fait, nous attendons avec une certaine impatience le livre blanc sur la défense qui doit être publié mercredi. Si la proposition de cessez le feu élaborée à Djeddah a légèrement fait bouger les lignes diplomatiques, et si des discussions techniques ont débuté aujourd’hui, la situation reste hautement préoccupante. Depuis le 11 mars, la position russe demeure largement ambiguë. Bien sûr, tout part du revirement des États Unis, la position de l’administration de M. Trump tranchant largement avec le soutien de son prédécesseur à l’Ukraine. Le rapprochement avec la Russie crée une instabilité manifeste, qui force l’Europe au réveil. Pour l’heure, beaucoup jugent la politique de Donald Trump erratique et peu compréhensible. Nous espérons qu’elle le soit, en fait, plutôt que d’imaginer que la stratégie actuelle est parfaitement pensée et voulue : cela ne la rendrait que plus dangereuse. En effet, la thèse selon laquelle les États Unis seraient en train de laisser le champ libre à la Russie sur le vieux continent devient de plus en plus plausible. plausible. Ce bouleversement que nous connaissons depuis quelques semaines, nous n’avons plus d’autre choix que de le comprendre comme une occasion offerte à l’Union européenne. Il sera, espérons le, l’électrochoc qu’il fallait à l’Europe pour qu’elle commence à réinvestir collectivement dans sa défense et dans sa souveraineté, sans compter aveuglément et sur le soutien des États Unis. 800 milliards d’euros qui devraient ainsi être mobilisés par la Commission européenne. Cette nouvelle donne n’en demeure pas moins catastrophique pour l’Ukraine. Cela fait un peu plus de trois ans que ce pays subit l’invasion russe, trois ans que les Ukrainiennes et les Ukrainiens s’épuisent à défendre leurs vies et leur territoire, face à un État russe toujours plus autoritaire. À l’issue du Conseil européen du 6 mars dernier, tous les États membres de l’Union, à l’exception notable de la Hongrie, ont réaffirmé les conditions indispensables à la paix entre l’Ukraine et la Russie : une paix globale, juste et durable, des négociations qui incluent nécessairement l’Ukraine et l’Europe et surtout, une paix qui respecte l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. À la différence du président et du vice président des États Unis, membres éminents de l’internationale réactionnaire, nous ne voulons pas d’une paix au rabais, impliquant une répartition des territoires et des ressources ukrainiens. D’ailleurs, de leur côté, les États Unis semblent parfois hésiter. Ils cessent les livraisons d’armes et de renseignements un jour pour les reprendre le lendemain… La seule conclusion que nous pouvons tirer de cette séquence est que les États Unis ne sont plus un allié fiable. L’Europe doit en tirer les conséquences. Une série de questions se pose, aussi, d’un point de vue financier. Pouvons nous à la fois maîtriser nos déficits publics, dépenser davantage pour nos armées respectives et accélérer notre soutien à l’Ukraine ? La réponse est non.

également, Donald Trump tente de rebattre les cartes pour montrer au monde entier ses talents de. Mais la diplomatie, la bonne diplomatie, s’improvise rarement, surtout lorsque les propositions formulées sont aberrantes, à l’instar de cette idée de transformer Gaza en Riviera du Proche Orient. Le groupe du RDSE ne peut qu’affirmer l’absolue nécessité de respecter le droit international et les droits fondamentaux des individus. L’Union européenne et la France doivent peser de tout leur poids pour que le cessez le feu actuel entre le Hamas et Israël et les échanges de prisonniers et d’otages se poursuivent dans de bonnes conditions, afin que le cessez le feu temporaire devienne définitif. Qu’il s’agisse de l’Ukraine ou du Proche Orient, l’enjeu pour l’Europe et pour la France n’est pas simplement de mettre un terme aux conflits, qui ne cessent de se multiplier et de prendre de l’ampleur ; il est d’établir les conditions d’une paix juste et durable entre tous les belligérants. La parole

On croyait l’Union incapable de recourir à l’endettement commun, jusqu’à ce qu’une pandémie l’y contraigne. On la pensait figée dans ses dépendances, jusqu’à ce que l’invasion de l’Ukraine par la Russie impose un tournant majeur. Aujourd’hui, l’Europe doit impérativement renforcer son autonomie stratégique. Cela passe par le rehaussement de nos dépenses militaires, mais aussi par un investissement massif dans notre souveraineté économique et technologique, afin de soutenir à la fois la réindustrialisation du continent et la transition écologique. Dans le domaine de la défense, il y a une première évidence : nous devons instaurer une préférence européenne dans les achats militaires. Mais la question centrale demeure bien entendu le financement de l’effort. La présidente de la Commission a annoncé a annoncé un plan de 800 milliards d’euros pour la défense européenne, dont 150 milliards d’euros seraient mutualisés un prêt européen, le reste reposant sur les dépenses individuelles de chaque État membre. Pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, cet effort ne saurait se traduire par des coupes budgétaires qui fragiliseraient notre modèle social. Il ne saurait non plus servir de prétexte pour enterrer toute modification de la réforme des retraites. d’éviter que cet effort ne se fasse au détriment de dépenses utiles à nos concitoyens, l’Union européenne devra également être capable de mobiliser

Autre conséquence de la nouvelle donne géopolitique : les cours boursiers des industries de défense connaissent un envol depuis plusieurs mois. Le risque de superprofits est bien réel. Quelles mesures sont envisagées pour éviter qu’une rente de situation ne se forme sur le chaos géopolitique ? Notre souveraineté ne se résume pas aux chars et aux canons. L’effort doit aussi porter sur les infrastructures numériques : réseaux sociaux, intelligence artificielle, cybersécurité, stockage et protection des données. L’Europe ne peut plus se contenter d’être un marché captif, en proie aux ingérences étrangères d’États qui cherchent à l’affaiblir. Reprendre la main passe par le développement de plateformes souveraines, financées par des fonds publics. Tel est notamment l’objet de la proposition de résolution européenne sur la

Enfin, notre quête de souveraineté ne doit pas se faire au détriment de nos engagements sociaux et environnementaux. La compétitivité et la simplification sont des enjeux clés, mais elles ne doivent pas servir de prétexte à un nivellement par le bas. Simplifier les normes Oui. Baisser le niveau d’exigence ? Non ! Quelle est la position de la France sur la révision des directives CSRD et CS3D, notamment sur la condition suspensive ? Monsieur le ministre, une Europe forte ne peut être qu’une Europe qui protège, qui régule et qui innove. La parole